la demande du groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, présentée par MM. Guislain Cambier, Jean Baptiste Blanc et plusieurs de leurs collègues

La loi, c’est ce sur quoi une société s’accorde pour déterminer son futur commun. La loi unit ; elle ne divise pas. Elle incarne une vision et fait l’objet d’un consensus. Hélas, parfois, ce n’est pas le cas. Nous pouvons le regretter. Notre rôle est surtout de corriger pour apaiser, rassembler les habitants et les projeter vers un avenir plus engageant. Nous le savons, l’artificialisation est une nécessité et un défi. Depuis l’aube de l’humanité, l’homme transforme son environnement. Il l’aménage. Nous avons glorifié les voies romaines, célébré les civilisations urbaines, réparti les espaces entre rural et urbain en fonction de leur rapport à la communauté. Parce que nous sommes les thuriféraires du progrès et non ses contempteurs, nous savons que la finalité, la nature et le nombre des aménagements évoluent. Nous devons donc poser une vision à long terme, sans nous enfermer dans des schémas. Nous devons rester pragmatiques. pour que la loi soit l’expression de la volonté générale, elle doit reposer sur un diagnostic partagé. Oui, nous avons artificialisé de manière peu économe dans les dernières décennies, poussés par un système financier et fiscal faisant de la terre une denrée de peu de valeur. Peut on continuer à ce rythme ? Non, car le sol, par nature, est précieux ; le protéger, c’est permettre à la population de bien vivre à l’avenir. Ce diagnostic, les élus et les acteurs le partagent. Les auditions, les réponses aux sondages que nous avons menés de manière transpartisane et constructive le démontrent. Mieux, elles prouvent que ces mêmes élus locaux et acteurs n’artificialisent qu’avec raison et parcimonie. Le changement est à l’œuvre ; il faut s’en féliciter, l’encourager et non le morigéner comme des doctrinaires ou des prescripteurs de morale. Nous vous proposons une loi de confiance, car responsabilité rime avec liberté, pas avec répression. Le discours de la méthode, c’est être rationnel et non passionnel. Sur les différentes travées de cet hémicycle, nous avons donc pris, ensemble, nos responsabilités. Pour aider les territoires dans leur diversité à construire eux mêmes le chemin du progrès, nous leur permettons de trouver ce difficile équilibre, ce chemin de crête, cette « trace » entre l’impérieuse nécessité de changer de modèle et la volonté inaliénable de se développer. Nous ne devons en exclure aucun. C’est cela, la promesse républicaine : garantir à chacun l’accès au progrès. Cette loi est un chemin, non un terminus. Qui serions nous pour édicter ce que seront la France et le monde en 2050 ? Gardons l’humilité propre à notre nature humaine. Ce passage étroit est guidé par le respect de chaque habitant, quel que soit l’endroit où il réside. Afin d’éviter qu’il ne trébuche sur ce chemin, nous voulons lui donner un cap clair, sans codicille. En temps de brouillard, comme de nos jours, les annexes obscures ne protègent que les initiés. Tremblons avant d’ajouter des exemptions, des références à des décrets ou à d’autres normes. Pour que tous les territoires puissent comprendre et appliquer la loi, il faut que celle ci soit claire. C’est dans la clarté que nous pouvons bâtir l’idéal de notre République, pas dans les obscurs bureaux d’une administration hors sol ! Mes chers collègues, nous vous proposons six articles. C’est peu, moins que le Décalogue…

Elle se veut surtout éclairante, aidante pour une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux (Trace). Cette Trace doit désormais remplacer un acronyme qui, malgré ses ambitions initiales méritoires, était devenu un repoussoir pour trop d’élus locaux. locaux. Mes chers collègues, ces six articles permettront tout simplement d’atteindre l’objectif partagé et nécessaire de la sobriété foncière : une comptabilité claire ; une trajectoire qui donne confiance ; un calendrier revu pour permettre une différenciation ; une conférence reposant sur le dialogue ; enfin, une territorialisation véritable. Aurons nous tout réglé ? Non. Il restera des chantiers à ouvrir sur l’équité territoriale, la ressource financière, la justice fiscale ou encore la santé des sols.

Le Parlement est une nouvelle fois appelé à légiférer sur la lutte contre l’artificialisation. Il le fait une nouvelle fois sur l’initiative du Sénat, qui, depuis quatre ans, tente de corriger les effets de la loi Climat et Résilience. Monsieur le ministre, voilà quatre ans que le Sénat se bat pour porter la voix des territoires, entre la condescendance de la haute administration, le mépris de certains préfets à l’égard de la volonté du législateur et les fausses pudeurs des gouvernements successifs vis à vis de l’écologie radicale. Peut être faudra t il écrire un jour l’histoire du zéro

S’est ensuivie la vassalisation des régions par l’État, trop heureux de pouvoir recentraliser à peu de frais l’aménagement du territoire et le développement urbain. Le mépris a continué avec les déclarations d’une ministre annonçant fièrement la fin du modèle pavillonnaire à tous ces Français qui avaient le malheur d’être enfin propriétaires. Je pourrais encore évoquer

opposabilité le moment venu. Le Sénat s’est donc une première fois mobilisé pour parer au plus urgent, en corrigeant les absurdités les plus manifestes du ZAN. C’est la loi de 2023, qui a permis de redonner un peu d’air aux élus, grâce notamment au droit à l’hectare. Nous savions qu’une grosse partie du travail restait à accomplir.

Avec nombre d’entre vous, mes chers collègues – je pense notamment à Guislain Cambier, à Jean Claude Anglars, à Amel Gacquerre et à Daniel Gueret –, nous avons considéré qu’il fallait traduire au sein d’une nouvelle proposition de loi les principales demandes de ces élus. C’est ce qui nous permet de vous présenter ce soir un texte légitimé par la signature de plus de 160 collègues.

de décider eux mêmes, en fonction des réalités locales, du rythme et de la pente de leur trajectoire de sobriété, grâce à un contrat – je dis bien : un contrat ! – qui prévoira toutes les clauses de rendez vous nécessaires. agricoles et forestiers (Enaf) après 2031 et laisser un peu plus de temps aux collectivités pour modifier leurs documents d’urbanisme. Nous faisons enfin le choix de renforcer le poids des communes au sein des conférences régionales.

votre expérience d’élu local nous conduit à beaucoup espérer de votre action. Votre regard bienveillant sur ce texte, malgré des désaccords qui persistent – c’est normal –, doit nous permettre d’avancer ensemble pour parvenir aux solutions les plus pertinentes, dans l’intérêt de la transition écologique. Celle ci passe nécessairement par l’accompagnement des élus. Je suis certain que vous aurez l’autorité nécessaire pour faire respecter un principe démocratique ancien. En 2025, l’administration doit obéir au pouvoir politique et à la volonté souveraine de la Nation que nous exprimons

voilà quasiment deux ans jour pour jour, le 16 mars 2023, le Sénat adoptait la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du zéro artificialisation nette au cœur des territoires, sur l’initiative de notre collègue Jean Baptiste Blanc. Ce texte a permis des avancées certaines sur le traitement des grands projets, une meilleure concertation à l’échelon régional et, surtout, la garantie de développement communal, essentielle pour les petites communes rurales. Malgré cela, deux ans plus tard, nous avons été obligés de remettre l’ouvrage sur le métier. Car, comme le pointait au mois d’octobre dernier le rapport du groupe de suivi sur l’artificialisation des sols, pour nos élus et pour nos collectivités, satisfaire aux obligations de réduction de l’artificialisation fixée par la loi Climat et résilience à droit constant relève véritablement de la quadrature du cercle. Dans toutes les réunions d’élus, le ZAN est le sujet numéro un ! Je remercie d’ailleurs l’ensemble de nos collègues, avec lesquels nous avons beaucoup échangé et qui nous ont aidés à prendre le pouls du terrain en temps réel. Je voudrais plus particulièrement remercier Guislain Cambier, président du groupe de suivi, et Jean Baptiste Blanc – j’ai assisté à beaucoup de réunions de ce groupe avec eux durant ces dernières années – d’avoir pris l’initiative de cette proposition de loi. Et je les félicite d’avoir effacé cet acronyme affreux de ZAN

Ce mode de comptabilisation est plus simple. Il a l’avantage de lever la contrainte sur les bâtiments agricoles. Dans ce cadre, la Commission a clarifié la notion de consommation d’Enaf, afin de donner aux élus davantage de visibilité sur la manière dont seront décomptées leurs consommations futures. L’article 5 imaginait une grande conférence régionale des maires pour débattre des enveloppes foncières. Par souci de stabilité, nous avons finalement conservé les conférences régionales de gouvernance mises en place en 2023, mais en augmentant la proportion des représentants des élus. La commission a également introduit un nouvel article qui aménage les modalités de mutualisation de la garantie de développement communal d’un hectare. Cette dernière a constitué une bouffée d’oxygène pour les communes rurales, qui étaient menacées par la loi Climat et Résilience de se voir privées de toute capacité de développement et d’être mises sous cloche. Mais les modalités d’application de cette garantie, élaborées dans l’urgence, aboutissaient dans certains territoires à des gels de foncier, préjudiciables pour d’autres collectivités. Ainsi, la mutualisation pourra

Enfin, la procédure de modification simplifiée pourra être utilisée pour inscrire concrètement dans les documents d’urbanisme les effets de cette garantie ou de sa mutualisation, y compris en cours de période.

est bon que l’on puisse laisser une trace de bon sens. Je voudrais remercier Amel Gacquerre de notre excellente collaboration sur un sujet sensible et techniquement difficile,

tenu à les associer constamment à nos réflexions, et ils se sont montrés ouverts aux évolutions que nous avons proposées sur ce texte. Je vous remercie également, monsieur le ministre, de votre écoute attentive et des échanges que nous avons d’ores et déjà pu

et je ne doute pas que cette proposition de loi pourra aboutir très prochainement. Le Gouvernement a d’ailleurs décidé d’engager la procédure accélérée sur ce texte, afin que celui ci puisse être adopté et entrer en vigueur avant l’été. C’est indispensable compte tenu des délais limites de modification des documents de planification et d’urbanisme actuellement en vigueur, ainsi que de la date des prochaines échéances électorales. Je souhaite également saluer l’engagement de nos collègues des différents groupes, qui ont, eux aussi, recherché le compromis. Je sais qu’ils l’ont fait dans un esprit de réalisme et de responsabilité, car ils constatent, comme nous, que la loi Climat et Résilience entraîne des blocages aux conséquences dommageables pour nos territoires. Si nous ne faisons rien, c’est toute une partie de la France périphérique, la France des campagnes, des bourgs et des sous préfectures, que nous risquons de perdre. C’est tout l’inverse ! Dans le cadre de l’examen de ce texte, nous avons cherché à être pragmatiques, en soutenant deux orientations. Premièrement, la politique de sobriété foncière ne doit pas être un frein à la mise en œuvre de toutes les autres politiques publiques. Bien entendu, 20 000 hectares artificialisés chaque année, c’est trop ! Nous aspirons tous à la préservation de nos terres agricoles de notre biodiversité. Mais il faut aussi prendre en compte la réalité de nos territoires. À ce jour, le foncier économique, par exemple, manque déjà. Deux tiers des intercommunalités ont déjà dû refuser des implantations d’usines par manque de foncier. Aggraver la situation n’est pas acceptable, notamment lorsque l’on met la réindustrialisation en tête de l’agenda politique. C’est une question de cohérence. C’est pourquoi, en commission, nous avons introduit des exemptions temporaires

de manière pragmatique, chacun à son rythme, et, surtout, en fonction des dynamiques territoriales. C’est pourquoi nous demandons aux régions, en concertation avec les conférences régionales d’élus, que nous avons renforcées, de se fixer elles mêmes une trajectoire permettant d’atteindre le zéro à à horizon 2050. Car ce sont les territoires qui sont les mieux à même de définir leur propre trajectoire, compte tenu de leurs contraintes, de leurs projets et de leurs besoins. Cette trajectoire devra être balisée par des objectifs intermédiaires chiffrés de réduction de la consommation foncière. Je dis bien des objectifs », c’est à dire au moins deux objectifs intermédiaires d’ici à 2050. Cela nous paraissait suffisant pour assurer la crédibilité de cette trajectoire. Pour autant, nous avons entendu les craintes d’une mise en œuvre du ZAN trop hétérogène, que certaines régions commenceraient trop tard. Nous vous proposerons donc, au nom de la commission des affaires économiques, un amendement tendant à fixer ce premier jalon à 2034

car les dynamiques ne sont pas les mêmes partout, et elles ne demeureront pas constantes d’ici à 2050. Les discussions se poursuivront, ce soir, demain, puis à l’Assemblée nationale, mais une chose est sûre : nous avons le devoir d’avancer ensemble pour faire aboutir ce texte, car il ne peut y y avoir de loi ZAN 4. S’il y a une nouvelle loi relative à l’objectif ZAN, elle devra porter sur les dispositions budgétaires et fiscales qui inciteront les élus à aller vers plus de sobriété foncière. La parole

pour la troisième fois en moins de quatre ans, nous voilà attelés à l’examen d’un texte ayant vocation à améliorer le cadre normatif de la sobriété foncière, faisant de ce sujet législatif un véritable travail de Pénélope. Depuis que la loi Climat et Résilience a instauré, dès le lendemain de sa promulgation et sans période transitoire, une trajectoire prescriptive et une méthode descendante pour atteindre des objectifs qu’il est permis sans exagération de qualifier d’ambitieux, tous les parlementaires sont devenus, bon gré mal gré, des pédagogues du ZAN dans les territoires. N’ayant pas été associés à la définition des cibles ni aux modalités pour y parvenir, les élus locaux ont bien souvent été perplexes, voire inquiets des conséquences de la mise en œuvre de cette stratégie en matière de développement local et d’attractivité. Pour comprendre les réticences relatives au changement de dimension de la sobriété foncière, il est préférable d’invoquer Descartes, plutôt que Montesquieu : c’est le discours de la méthode qui est perfectible et à revoir, et aucunement l’esprit de la loi, qui fait d’ailleurs l’objet d’un large consensus quant à ses finalités. Il existe en effet d’impérieux arguments scientifiques en faveur du renforcement des efforts en matière de sobriété foncière ; on pourrait même dire qu’il s’agit d’une ardente obligation. La gestion économe de l’espace n’est pas un luxe, non plus qu’une mode urbanistique ; c’est une nécessité dûment attestée par les études scientifiques, qui convergent toutes vers les mêmes constats. La préservation des sols se situe en effet à la convergence des trois principaux enjeux environnementaux : biodiversité, régulation du cycle de l’eau et atténuation climatique. Plus l’on protège les fonctions écologiques, meilleurs et plus efficaces sont les services écosystémiques rendus, tout en tout en maintenant leur potentiel agronomique., en adoptant une approche négative, les effets directs et indirects induits par la dégradation des sols coûtent de plus en plus chers à la société : inondations, pollution du fait d’un ruissellement accru des eaux, baisse de la capacité de stockage de CO2 et fragmentation des espaces naturels qui concourt à l’érosion de la biodiversité, etc. Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit à l’erreur : nous devons renforcer et sécuriser notre trajectoire vers la sobriété foncière, car il s’agit de la condition de la réussite de la transition écologique. Nous devons stabiliser le cadre normatif et mettre fin à l’insécurité juridique découlant de ce que le législateur n’a de cesse de remettre l’ouvrage sur le métier. C’est précisément l’objet et la raison d’être de la proposition de loi Trace : réussir la sobriété foncière en associant plus étroitement les élus locaux à la répartition territoriale des efforts. Ce fil rouge a guidé l’approche de la commission des affaires économiques et la nôtre, celle de l’aménagement du territoire et du développement durable. Elle a conduit à travailler en étroite collaboration, pour assouplir sans dénaturer. Dans le temps qui m’est imparti, je ne vous présenterai pas dans le détail les six articles de la proposition de loi, exercice auquel se sont brillamment livrés les rapporteurs au fond. J’insisterai simplement sur le fait que notre commission a confirmé son attachement à l’ambition originelle figurant dans la loi Climat et Résilience, à savoir réduire graduellement le rythme national des consommations foncières, pour atteindre l’absence d’artificialisation en 2050. Pour y parvenir, nous avons proposé, conjointement avec la commission des affaires économiques, des évolutions calibrées et des assouplissements encadrés permettant aux territoires de déterminer les trajectoires adaptées à leurs spécificités et à leur dynamisme, tout en veillant au réalisme du rythme fixé. Il s’agit d’un véritable acte de foi en la capacité des élus locaux de s’emparer de ces sujets et de promouvoir des modèles d’aménagement durable, plus sobres en foncier. Nous nous sommes efforcés d’introduire des dispositions de mise en cohérence de nos politiques publiques, en veillant par exemple à ce que l’État s’astreigne lui aussi à la même rigueur foncière, en conservant la comptabilisation en Enaf, en évitant que la stratégie de sobriété foncière ne fasse obstacle à la réindustrialisation et à la relocalisation des activités souveraines, en reportant les dates butoirs de modification des documents d’urbanisme, en faisant évoluer les modalités de mutualisation de mutualisation de la surface minimale dont bénéficient les communes, tout en instaurant un dialogue territorial qui permet tout à la fois d’associer les élus et d’assurer la capacité décisionnaire de la conférence régionale. c’est en partant des territoires et en associant plus étroitement les élus locaux à la définition des cibles intermédiaires et à la territorialisation des objectifs que la sobriété foncière deviendra un objectif commun et partagé, et non plus une stratégie qui exaspère les collectivités,

je souhaite que nous puissions ensemble tracer, si vous me permettez ce jeu de mots, le chemin vers un ZAN qui soit compris dans ses ambitions et assoupli dans ses conditions de mise en œuvre. Mon objectif est de rassurer l’ensemble des élus locaux sur l’adéquation de cet objectif avec la poursuite de stratégies d’aménagement du territoire durables et équilibrées.

parfois de manière ambitieuse, dans la mise en œuvre du ZAN. Je le dis depuis le début, je considère qu’il faut repartir des territoires non pas d’imposer depuis Paris, mais bien de bâtir des solutions adaptées aux réalités, que vous connaissez tous, de chaque territoire. La discussion s’engage donc autour de ce texte, dont l’objectif vous l’avez rappelé à plusieurs reprises – est non pas de supprimer le ZAN, mais de construire ensemble une trajectoire pour honorer notre objectif de 2050. Le cap est fixé ; il n’a pas varié. Les ajustements que vous suggérez ou que je proposerai permettront sans doute de mieux s’y préparer, mais nous devons veiller à ce que la trajectoire soit respectée, car elle est fondamentale, je le crois, pour l’avenir de notre pays. C’est un point sur lequel je reviendrai.

Vous le savez, l’étalement urbain pénalise nos centres villes, accroît notre dépendance aux mobilités carbonées, éloigne nos concitoyens de l’accès aux services et aux équipements publics, et parfois même de l’emploi.

pour 21 % des nouveaux habitants et 29 % des nouveaux ménages. Le déséquilibre peut s’entendre au regard de la nécessité de pallier les difficultés réelles liées à l’isolement, mais nous ne pouvons nous satisfaire pleinement

entre les territoires, laissant certaines zones rurales et urbaines enclavées ou délaissées. Nous devons donc œuvrer contre l’éparpillement des activités et la désertification des cœurs de ville, en faveur de la cohésion et contre l’émiettement d’une part de notre tissu social et de l’attractivité économique des territoires. Or, chaque année,

que je lancerai prochainement avec mes collègues Éric Lombard et Agnès Pannier Runacher. Il me paraît judicieux de prévoir de s’appuyer sur ses conclusions

en retard d’atteindre l’objectif en 2050. Il s’agit non pas de pointer du doigt ou de mettre en jugement les collectivités qui n’arriveraient pas à tenir cet objectif, qui pourra d’ailleurs s’apprécier avec discernement,

C’est ainsi que je vous proposerai, en accord avec mon collègue Marc Ferracci, un dispositif dédié à ces implantations industrielles.

Ainsi, à compter de la date de promulgation de la présente loi, les projets industriels auront vocation à émarger prioritairement sur cette enveloppe, plutôt que sur l’enveloppe des Pene. Cette réserve, dont la consommation foncière

En outre, l’inscription des projets dans l’enveloppe nationale dédiée à l’industrie se fera selon une procédure simple et concomitante au dépôt des autorisations d’urbanisme.

par décret en Conseil d’État. Enfin, pour garantir la transparence de l’action publique, la liste de ces projets sera rendue publique. Par ailleurs, je partage la nécessité de revenir à une méthode de comptabilisation en

elle conduit à renoncer à une appréciation plus fine des dynamiques d’occupation et d’usage des sols. Je n’ai pas déposé d’amendement, afin de permettre la discussion autour de vos propositions, mais je rejoins les rapporteurs sur ce point. Je tiens par

je suis favorable à l’inscription dans la loi d’une forme de définition des zones périurbanisées, afin de traiter, notamment, des dents creuses. Pour ne pas rigidifier le dispositif permettre une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, je propose de nous appuyer sur la notion de faisceau d’indices, issue de la jurisprudence. Cette différence de comptabilisation ne doit cependant pas altérer la définition de l’artificialisation ; j’y reviendrai. J’entends également votre souhait de vous appuyer sur les conférences régionales de gouvernance, que vous avez lancées, pour replacer les élus locaux au cœur des stratégies territoriales d’atteinte du ZAN.

à ce que ces assouplissements n’aient pas un effet contre productif, qui pourrait nous éloigner de l’objectif à horizon 2050. Aussi, le compromis que je propose – décaler la période d’observation à 2034 entraînera un assouplissement de la trajectoire d’environ 37 500 hectares, avec l’exemption des grands projets industriels, en faisant porter ces 10 000 hectares sur ce volume de 37 500

Cependant, certaines d’entre elles, tout comme les propositions qui vont nourrir le débat, présentent à mon sens un risque important de vider de leur substance les engagements auxquels nous sommes attachés.

ne pouvaient pas réellement maîtriser – cela semble aujourd’hui évident – leur consommation foncière. Je le redis, ma proposition permet de détendre l’objectif initial de 37 500 hectares, qui pourront donc être mobilisés par les collectivités

En effet, il est nécessaire que l’évolution des documents d’urbanisme ait lieu pendant la période d’observation, afin de donner aux collectivités les moyens d’ajuster leur stratégie et de mettre en œuvre les orientations inscrites dans leur document d’urbanisme pendant cette période.

ces trois lettres que nous avons tous identifiées continuent de susciter tantôt des critiques, tantôt des inquiétudes, parmi les élus locaux de France. Si nous pouvons avoir le sentiment que ce concept existe depuis de nombreuses années, il fut un temps, pas si lointain, où nous parlions du sujet de l’artificialisation sans faire référence au ZAN. En réalité, mes chers collègues, la notion est apparue en 2018, à l’occasion du plan biodiversité lancé par le ministre Nicolas Hulot. La notion fut ensuite reprise par la Convention citoyenne sur le climat, face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, qui fixa l’objectif zéro artificialisation nette pour 2025. Sur le papier, l’intention était louable, mais force est de constater que sa mise en place a été chaotique pour les élus. Entre le manque de concertation avec les principaux acteurs concernés et des méthodes de comptabilisation plus que complexes, le ZAN s’est heurté à la réalité de nos territoires. Sans oublier la publication de décrets qui ne correspondaient pas à la lettre de la loi Climat et Résilience, ce qui n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres…

Cette loi a certes apporté des assouplissements, mais sans lever pour autant tous les blocages. C’est la raison pour laquelle le Sénat a décidé de lancer un groupe de suivi des dispositions législatives et Ce groupe de suivi, dont j’ai été membre, avait lancé en 2024 une concertation en ligne à destination des élus locaux. Les résultats, publiés en juin 2024, sont sans appel 75 % des répondants estiment que les critères de territorialisation des enveloppes d’artificialisation ne sont pas correctement pris en compte ; 77 % des répondants bénéficiaires de la garantie de développement communal ont l’intention de l’utiliser plus des deux tiers des répondants ont du mal à déterminer ce qui est classé comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ; enfin, 81 % des répondants considèrent le changement de mode de comptabilisation de l’artificialisation en 2031 comme problématique… Autant de raisons qui justifient, mes chers collègues, de réajuster le ZAN. Tel est le sens de cette proposition de loi : repenser le ZAN pour en faire un outil intelligent et adapté aux réalités locales. Plutôt que d’avoir une logique verticale et descendante, je crois qu’il serait bénéfique pour tout le monde d’inverser la logique de territorialisation, en partant des besoins et des projets des collectivités territoriales. Je trouve donc utile de pérenniser, au sein de l’article 1, la mesure de l’artificialisation par le décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les Enaf, comme c’est actuellement le cas jusqu’en 2031. Ce mode de comptabilisation, connu et compris des élus locaux, permet aux collectivités de mieux piloter leur artificialisation au travers de leurs documents d’urbanisme et d’assurer un suivi en temps quasiment réel des consommations foncières. discussion du mode de calcul est justement l’occasion de réfléchir à la nature même des projets inclus dans la comptabilisation, laquelle fait régulièrement l’objet d’interpellations de la part de nos maires. À ce propos, je salue l’adoption d’un sous amendement que j’ai défendu en commission et dont le but est d’exempter du décompte de la consommation d’Enaf les énergies renouvelables jusqu’en 2036. En effet, la décarbonation du mix énergétique et la sobriété foncière ont les mêmes objectifs : lutter contre le dérèglement climatique et renforcer notre souveraineté énergétique. La mesure a été adoptée en commission – tant mieux Nos débats en commission ont également démontré la nécessité de revenir sur les dates butoirs s’agissant des documents d’urbanisme. En ce sens, le décalage de ces dates me semble bienvenu. Concrètement, il s’agit de repousser les dates butoirs de 2027 et 2028 avant lesquelles doit intervenir la modification des documents d’urbanisme, à 2031 pour les Scot et à 2036 pour les PLUi et les cartes communales. J’ajoute que les régions pourront, en toute souplesse, décider ou non de modifier leur Sraddet, afin d’adopter un objectif régional de trajectoire foncière jusqu’au 22 août 2026. Mes chers collègues, en conclusion, je crois que le Sénat peut, une fois encore, être la vigie attentive et soucieuse du quotidien des élus locaux. Il s’agit non pas de remettre en cause l’idée même du ZAN, mais simplement d’en faire un outil plus affûté, plus utile et plus adapté aux réalités locales. C’est une nouvelle occasion de prouver le sérieux de notre assemblée et, ainsi, de démontrer que la démocratie représentative est bel et bien utile dans notre pays. La parole

années ont suffi pour artificialiser davantage de terres qu’en cinq siècles. Ainsi, en Loire Atlantique, on a consommé autant de terres en un siècle et demi que depuis les origines de l’humanité Pour enrayer cette fulgurante accélération, la loi Climat et Résilience de 2021 a introduit l’objectif zéro artificialisation nette à horizon 2050. J’avais moi

: « N’attendez pas qu’une loi vienne vous dicter ce que vous devez faire. » J’étais, hélas ! visionnaire, tant cette loi a suscité rejet et défiance de la part de nos élus locaux. du dispositif, la parole peu ou pas écoutée des acteurs de terrain et les inégales interprétations des services décentralisés de l’État ont transformé un impératif de sobriété foncière en une entrave supplémentaire dans la gestion et le développement de nos territoires. Dès 2023, le législateur, ayant conscience de ces difficultés, y avait apporté des modifications la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte renforcer l’accompagnement des élus locaux, notamment autour des projets d’envergure nationale ou européenne, les Pene, par l’instauration de la garantie rurale et l’installation des conférences régionales. Néanmoins, cette initiative parlementaire bienvenue ainsi que les changements réglementaires qui ont suivi n’ont pas suffi à corriger tous les défauts d’un objectif initial mal conçu. Comment, dès lors, concilier sobriété foncière et développement du territoire, ces objectifs aujourd’hui compris et intégrés Il s’agit de trouver un point d’équilibre entre l’impératif moral de maintenir l’objectif ZAN pour garantir une terre vivable pour nos petits enfants, l’absolue nécessité d’assurer un logement pour tous et de garantir les conditions de notre souveraineté industrielle, si cruciale actuellement, et la prise en compte des diversités et des différents besoins de nos territoires. Dans ce contexte, le groupe RDSE aborde plutôt favorablement la discussion des articles 1, 3, 4, 5 et 6, qui redonnent de la capacité aux élus locaux en assouplissant la définition de l’artificialisation, en les libérant des fortes contraintes calendaires autour des documents d’urbanisme, ou encore en renforçant le rôle de la conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière. En revanche, nous estimons que l’article 2, qui vise à supprimer l’objectif intermédiaire, aujourd’hui fixé à 2031, n’est en aucune façon en aucune façon une mesure de souplesse, mais constitue au contraire une perte de repères. Le marin que je suis sait combien les balises sont indispensables pour atteindre le port sans encombre quand la mer est mauvaise… Sans balise intermédiaire, sans point d’étape, nous plongeons nos collectivités dans le brouillard et nous prenons le risque d’une aggravation des disparités territoriales.

n’est que le sillage que nous laissons derrière nous ; elle ne définit pas le chemin qui reste à parcourir ! Sans aucun point d’étape d’ici à 2050, comment ne pas craindre que certaines collectivités soient tentées de se mettre à la cape ? Quel héritage allons nous léguer aux maires qui seront élus en 2044 ? D’autant que – nous le savons, car le ministre l’a dit – les dernières marches pour atteindre l’objectif ZAN seront les plus difficiles à gravir. Comment nous jugeront ils alors ? Par conséquent, le Sénat doit assumer pleinement son rôle de chambre des collectivités et répondre aux attentes de nos élus : maintenir un objectif très ambitieux, pour laisser une terre désirable aux générations à venir sans pour autant imposer des contraintes obérant leur pouvoir d’agir rendre l’objectif ZAN soutenable sans le vider de sa substance ou, comme je l’ai répété tout au long de nos débats, ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain fixer le cap, tracer la route, pour que chaque commune de France puisse dessiner sa trace et l’inscrire dans son livre de bord. Voilà, mes chers collègues, ce à quoi je nous invite. La parole est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

L’application uniforme de ce dispositif issu de la loi Climat et Résilience s’est avérée profondément inadaptée aux réalités et aux besoins de ces derniers.

Nos élus se retrouvent trop souvent contraints, voire bloqués dans le développement de leur offre de logements ou d’accueil d’entreprises, alors même que nous prônons la réindustrialisation de notre pays

Mais il reste du chemin à faire. Je salue le travail de nos deux collègues auteurs de la proposition de loi et des trois rapporteurs, qui dressent le même constat.

Nous devons renforcer les moyens d’action pour accéder à la sobriété foncière et amoindrir une coercition contre productive. Il faut octroyer davantage de libertés aux élus, seuls à même de connaître les enjeux et les besoins en termes d’aménagement de leurs territoires. La différenciation territoriale sera un gage d’acceptabilité et d’adhésion.

d’urbanisme et le calendrier permettant aux conférences régionales de sobriété foncière de fixer les objectifs intermédiaires, ainsi que la conférence régionale du ZAN. réalisme puisque les projets industriels et les logements sociaux ne seront pas comptabilisés jusqu’en 2036. Voilà une vraie réponse aux attentes des territoires. La gestion des friches constitue un autre enjeu essentiel. Pour faire face à la désindustrialisation, il faut aider à la renaturation.

je souhaite ardemment qu’elle soit examinée au plus vite à l’Assemblée nationale pour permettre à nos territoires de tracer leurs projets sur le chemin du bon sens et des libertés locales. La parole

immédiatement que de nombreuses collectivités font l’effort de réduire leur consommation de foncier, en densifiant quand c’est possible ou en renaturant l’espace public dans les zones les plus bétonnées.

Comme nous, les maires souhaitent trouver un équilibre entre, d’une part, la préservation de la qualité de vie, celle de la biodiversité, des espaces naturels, agricoles et forestiers indispensables à la lutte contre le dérèglement climatique et, d’autre part, l’attractivité et le dynamisme de leur territoire, qui attirent et facilitent l’activité humaine. Nous devrons, demain, accueillir des équipements publics, construire des écoles tout en ayant des îlots de fraîcheur pour nos enfants. Nous devrons cultiver des terres agricoles, augmenter le nombre de surfaces et diversifier nos cultures, tout en accueillant des commerces. Nous devrons aussi réindustrialiser pour réduire nos émissions et ne pas consommer de produits conçus à l’autre bout de la planète, tout en évitant de délocaliser

C’est le cas de certains projets d’envergure nationale ou européenne, qu’il était important d’intégrer dans notre réflexion pour que la loi en tienne compte.

C’est aussi pour répondre à cette équation que nous avons de nouveau souhaité aborder la question des friches. Ces espaces bâtis, mais délaissés, nuisent à la fois aux objectifs de réduction de l’artificialisation et à l’attractivité de nos territoires. Nous aurions donc tout intérêt à renforcer leur traitement.

du temps et de la souplesse pour que tous atteignent leur objectif. C’est cette volonté qui a guidé les travaux du groupe de suivi dont est issue cette proposition de loi ; notre groupe en suivra la trace dans son vote final.

Nous jugeons que la proposition de loi Trace, en l’état, n’offre pas toutes les garanties nécessaires à la préservation des terres agricoles. Nous demandons donc que la proposition de loi soit retravaillée pour conserver des objectifs et des moyens ambitieux de préservation des terres agricoles.

! Pour ne pas laisser le pauvre Wauquiez seul face à ses surenchères populistes, il fallait que cet hémicycle lui même lui redonne une légitimité en soutenant sa position.

de remise en cause de la lutte contre l’artificialisation ? La non prise en compte de l’importance de la préservation des terres agricoles pour la souveraineté alimentaire, … Non ! … le refus de l’urgence de l’adaptation au changement climatique, alors que les espaces naturels et agricoles sont au cœur de la lutte contre les inondations. C’est un cadeau

la réduction de moitié de l’artificialisation dans les années 2030 et le zéro artificialisation nette à l’échelle nationale en 2050. Pour le groupe socialiste, la marche à suivre était claire dès le début et nous n’en avons jamais dévié. Dès 2021, nous soulignions la nécessité de territorialiser la mise en œuvre objectifs et demandions au Gouvernement de la lisibilité, une concertation ascendante, une égalité de traitement entre les territoires et, surtout, des moyens d’accompagnement. Or, quatre ans et deux propositions de loi plus tard, force est de constater que les blocages demeurent. Il y eut d’abord la loi d’initiative sénatoriale du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer Ce bel exemple de travail transpartisan, voté à l’unanimité par le groupe socialiste, avait déjà apporté des assouplissements : report des dates pour adapter les documents d’urbanisme, précision des critères de territorialisation, mutualisation à l’échelon national de l’enveloppe des Pene, prise en compte des friches.

entre les régions qui ont respecté la trajectoire, celles qui devront remettre l’ouvrage sur le métier et celles qui n’ont pas encore avancé, sans jauge permettant de vérifier si l’objectif est bien respecté Nous ne pouvons accepter ce texte en l’état. Nos amendements s’emploieront donc à rétablir certaines dispositions que nous estimons indispensables. Nous souhaitons un objectif intermédiaire commun de 50 % de réduction de terres artificialisées. Nous ferons différentes propositions en termes de jalons, afin de permettre aux territoires d’avancer à leur rythme.

Dans un souci de cohérence, nous avons également déposé un amendement visant à ne pas obliger les régions ayant déjà modifié leur document de planification à faire évoluer celui ci de nouveau. Comme en 2023, nous proposons de nouveau d’expérimenter un dispositif de pondération au bénéfice des projets ne conduisant Suivant l’idée de territorialisation que nous préconisons depuis quatre ans, cette mesure permettrait également de mieux intégrer la préservation des sols dans les politiques d’aménagement.

pour le suivi du foncier, ce qui constitue une mesure de simplification cohérente. Nous proposerons aux collectivités d’expérimenter un outil de diagnostic de la qualité et de la santé des sols, afin de les aider à mieux orienter leurs choix urbanistiques en ciblant l’artificialisation sur des sols aux performances agronomiques moindres, préservant ainsi les sols à fort potentiel. Toujours dans la perspective d’aider les communes déjà engagées dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière, nous souhaitons encourager les projets favorables à la neutralité climatique, afin que la territorialisation des enveloppes foncières n’empêche pas les communes de réaliser des projets favorisant la transition écologique. Enfin, nous formulerons une proposition concernant la garantie rurale de 1 hectare, qui a rapidement été dévoyée. Nous avions déjà demandé au Gouvernement de l’époque des garanties sur la mise en œuvre de ce dispositif, dont tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître la complexité. Il rend l’application de certains critères de territorialisation difficile et entraîne parfois un gel du foncier, soit l’inverse de l’objectif visé. Nous proposons donc une clause de revoyure, au plus tard en 2028, pour vérifier sa bonne articulation avec le dispositif de mutualisation et son incidence sur l’enveloppe foncière. Mes chers collègues, la ligne du groupe socialiste est claire et n’a pas changé depuis 2021 : nous sommes favorables à l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050, mais estimons nécessaire de définir un objectif intermédiaire et surtout de sanctuariser le travail déjà accompli par les collectivités territoriales. Il faut conclure ! J’espère que nos débats sauront être sereins, constructifs et intelligents, ce qui est le propre des débats du Sénat. Voilà qui apporterait un salutaire réconfort dans les temps politiques que nous vivons.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur une proposition de loi qui marque une avancée importante pour nos élus locaux. Trop souvent, ces derniers sont considérés comme de simples exécutants de décisions prises à Paris, sans qu’on leur laisse réellement la possibilité d’adapter les règles aux réalités de leur territoire. Or qui mieux qu’un maire sait comment gérer l’urbanisation de sa commune ? Qui mieux qu’un élu de terrain peut juger des besoins de sa population en matière de logement, de services ou de développement économique ? Ce texte permet enfin de remettre un peu de bon sens dans notre politique d’aménagement du territoire. Il prévoit une trajectoire plus réaliste et concertée de réduction de l’artificialisation des sols, en associant enfin les élus locaux aux décisions. Il clarifie des définitions floues, qui avaient jusqu’ici mené à des blocages injustifiés. En cela, il répond aux nombreuses inquiétudes soulevées par les maires et les élus municipaux qui, depuis la loi Climat et Résilience, se retrouvent piégés par des règles incohérentes et inapplicables. Le Rassemblement national soutient donc cette proposition de loi, car elle va dans le bon sens : celui d’un urbanisme équilibré, qui protège nos terres agricoles et naturelles tout en permettant aux communes de se développer harmonieusement. Depuis longtemps, Marine Le Pen alerte sur les conséquences absurdes des politiques écologistes punitives imposées par la technocratie parisienne. Nous l’avons dit et répété : la loi Climat et Résilience, telle qu’elle a été pensée, est une machine à empêcher, qui bloque la construction de logements, asphyxie les communes rurales et renforce les fractures territoriales. Cette proposition de loi corrige certaines erreurs et offre une bouffée d’oxygène aux collectivités. Mais nous devons rester lucides : si elle constitue une avancée, elle ne règle pas tout. Nous le savons, derrière sa volonté affichée de concertation, le Gouvernement poursuit sa politique de régionalisation à marche forcée. Nous devons ici le dire clairement : la logique de transfert de compétences aux régions se fait au détriment des petites communes. Le risque est évident : la centralisation se déplace non plus vers l’État, mais vers les métropoles, qui concentrent toujours plus de pouvoirs, de ressources et de décisions. À terme, ce sont encore nos villages et nos territoires ruraux qui en paieront le prix fort. Ce que nous voulons, nous, c’est que les communes, grandes ou petites, aient réellement les moyens de décider de leur avenir tout en gardant un contrôle foncier, afin de protéger les terres agricoles. Nous serons vigilants, car nous savons que l’avenir de nos territoires ne doit pas être dicté par des logiques bureaucratiques et technocratiques. Nous devons redonner aux maires la liberté d’agir, la liberté de construire et la liberté d’aménager leur territoire en fonction des réalités locales. Le combat du Rassemblement national est celui de la proximité, de la souveraineté locale et du respect des élus, qui œuvrent au quotidien pour leurs concitoyens. Cette proposition de loi va dans le bon sens, mais elle ne suffira pas à inverser la tendance si nous ne remettons pas en cause les grandes orientations imposées par le Gouvernement. Parce que nous croyons en la France des territoires, nous voterons pour ce texte proposé par les sénateurs Guislain Cambier et Jean Baptiste Blanc, mais nous continuerons de défendre une véritable politique d’aménagement du territoire qui ne sacrifie pas nos communes rurales et qui garantisse une réelle équité entre tous les Français, qu’ils vivent en ville ou à la campagne. La parole est à M. Cédric Chevalier. Monsieur le président,

Très bien ! Des contraintes frappent certains territoires, en particulier en ruralité. Une application uniforme crée des incohérences entre les territoires ruraux et les pôles urbanisés, qui ont la possibilité de reconstruire sur des En parallèle, et paradoxalement, notre pays doit répondre à des enjeux cruciaux – réindustrialisation, construction de logements, renforcement de notre souveraineté alimentaire et énergétique – qui peuvent donner lieu à de la consommation foncière. Or, face à ces nécessités, les rigidités imposées par la loi de 2021 rendent toute évolution extrêmement complexe. Il ne s’agit pas non plus de tomber dans l’excès inverse et d’être trop permissif : nous devons trouver le juste équilibre. Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec les élus locaux, seuls à même de construire un projet pour leur territoire tout en intégrant les grands enjeux de préservation des ressources naturelles. Ils sont en première ligne et constituent les meilleurs relais vis à vis de ceux de nos concitoyens qui seront affectés. Il faudra de la conviction et du dialogue pour expliquer à une famille ayant payé des droits de succession sur un terrain à bâtir que celui ci n’est plus constructible à cause du ZAN : bon courage !

C’est aussi l’occasion de leur redonner du temps, élément essentiel pour faciliter la réflexion, la projection et l’acceptation.

force est de le constater, presque quatre ans après l’adoption de la loi Climat et Résilience, l’inquiétude des élus locaux ne faiblit pas – bien au contraire – et l’application de cette loi devenue un enjeu central pour la compétitivité et la réindustrialisation de notre pays. Les assouplissements permis par loi du 20 dont je salue l’initiateur, Jean Baptiste Blanc, n’ont pas été suffisants pour assurer une application apaisée de cette politique, dont nous partageons pourtant tous la philosophie générale. Le groupe de suivi des dispositions

de l’aménagement du territoire ou des services publics, chaque audition nous a fourni de nouveaux témoignages sur les difficultés causées par cette politique de réduction de l’artificialisation. À cette situation, la proposition de loi de nos collègues Guislain Cambier et Jean Baptiste Blanc apporte deux réponses structurantes : elle fait sauter le verrou verrou de la réduction de 50 % de l’artificialisation des sols à l’horizon de 2031 et elle renforce le rôle des collectivités dans la définition des enveloppes foncières, à rebours de la logique descendante qui prévaut aujourd’hui.

Faire confiance aux territoires pour déterminer les meilleurs moyens d’atteindre l’objectif de zéro consommation nette d’espace en 2050 constitue bien évidemment la meilleure solution, une solution qui devrait transcender tous les groupes politiques. C’est aussi dans cet esprit transpartisan que la majorité sénatoriale a constamment refusé depuis 2021 de remettre en cause l’objectif de neutralité foncière en 2050. Cette proposition de loi ne fait pas exception : pas un seul amendement n’a été déposé en ce sens. Toutefois, le ZAN ne saurait signifier « zéro avenir net » pour notre industrie, pour la ruralité et tout simplement pour notre pays.

tous nous le disent, du patron de PMI au dirigeant de grand groupe : le manque de foncier est un problème majeur pour l’attractivité de notre pays. Absolument ! Sortir l’industrie de la comptabilisation ne relève donc pas d’une lubie, c’est la réponse à un problème structurel, qui grève notre compétitivité. Enfin, nous sommes particulièrement attentifs à ce que la politique de sobriété foncière n’affecte pas de manière disproportionnée nos territoires ruraux, qui ont souvent été vertueux par le passé. La garantie de développement communal matérialise un « droit au projet » essentiel pour chaque commune : ses aménagements, qui rendent le dispositif plus opérationnel et permettent d’assurer sa pérennisation, sont tout à fait bienvenus,

grâce auxquels, du fait de l’engagement de la procédure accélérée, nous pouvons envisager l’adoption définitive de ce texte avant la fin de la session. J’y vois la confirmation qu’il est possible, dans le contexte politique que nous connaissons, sur le fondement d’une initiative et d’un travail approfondi du Sénat, de créer une majorité de projet autour d’un texte structurant pour l’avenir de notre pays. C’est la voie de la responsabilité, celle que le groupe Les Républicains a choisie ; soyons toujours plus nombreux à suivre cette trace là

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà de nouveau rassemblés pour aborder un sujet qui n’en finit pas de cristalliser les tensions chez les élus : l’usine à gaz qu’est La simplification est un thème qui me tient à cœur : simplification des normes pour nos entreprises, mais aussi simplification pour nos élus et nos concitoyens. La proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux s’inscrit totalement dans cette démarche. Un aménagement durable plus économe en foncier est bien évidemment capital, mais nous ne devons pas pour autant altérer les dynamiques de nos territoires, que celles ci soient liées à l’habitat ou au développement économique.

Aujourd’hui, personne ne souhaite les récupérer et les renaturer. Les retraités agricoles ne peuvent financer la renaturation avec leurs petites pensions et est ce vraiment rendre service à un jeune agriculteur que de lui transmettre un bâtiment amianté à réhabiliter ?

un très grand nombre de ces hameaux ne sont pas considérés comme des secteurs déjà urbanisés, ce qui obère la possibilité de construire dans les dents creuses qui s’y trouvent. vous en conviendrez, il serait bien plus logique de densifier l’existant que d’étendre les limites de l’urbanisation. Pour ce faire, il nous faut prendre en compte les particularités de chaque territoire. la présente proposition de loi s’inscrit dans cette dynamique, en permettant la territorialisation des décisions plus importantes. Pour ces raisons et pour celles qu’a évoquées mon collègue Franck Menonville, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte. La

à l’automne dernier, trois de nos commissions permanentes étaient réunies pour adopter, dans un élan quasi œcuménique, le rapport d’information issu des travaux du groupe de suivi transpartisan sur la mise en œuvre du ZAN.

à l’aube de l’examen de cette proposition de loi dite Trace, nos sentiments oscillent entre une déception latente, des regrets face à des manques criants et une inquiétude majeure. Une déception, disais je, car, en dépit de l’étendue et de la richesse des auditions menées par le groupe de suivi, nous ne retrouvons pas dans cette proposition de loi l’exhaustivité des constats réalisés et surtout des préconisations émises en conclusion de nos travaux. Très juste ! Ces préconisations ne manquent pourtant pas et elles permettraient d’embrasser toutes les facettes du ZAN, ses limites comme ses opportunités.

Or une ingénierie digne de ce nom ne pourra voir le jour sans la massification de l’accompagnement des collectivités, notamment rurales, ce qui passera nécessairement par le renforcement des services déconcentrés de l’État

En légiférant dans ce sens, nous risquons d’ouvrir une boîte de Pandore juridique, dans laquelle les conflits interprétatifs seront légion et dont les élus locaux seront assurément les premières victimes. Il s’agit là de l’une des nombreuses limites évoquées il y a quelques instants par notre collègue Christian Redon Sarrazy.

est de porter une vision durable de l’aménagement du territoire national, fondée sur la cohésion entre les villes et les campagnes, la sobriété dans l’usage des sols et l’audace d’une transition écologique ambitieuse. Hélas ! à ce stade,

Son constat est clair : la mise en œuvre du ZAN est jugée trop rigide, trop technocratique et déconnectée des réalités locales. Placés en première ligne, les maires éprouvent des difficultés face face à l’accumulation de normes et à la rigidité des objectifs fixés sans réelle étude d’impact. Le ZAN est perçu comme une réforme technocratique imposée verticalement. Pis, certaines communes vertueuses, ayant déjà limité leur consommation foncière, se trouvent aujourd’hui pénalisées, d’où un sentiment d’injustice.

Ensuite, elle supprime l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation des sols d’ici à 2031, tout en maintenant celui de 2050. Toutefois, sans modification de la période de référence pour établir les objectifs de réduction, fixée à 2011 2021, l’effet de cette suppression restera limité. La réévaluation de cette base aurait été nécessaire pour mieux prendre en compte l’évolution des dynamiques territoriales. elle reporte également les dates butoirs de mise à jour des documents d’urbanisme, offrant une respiration bienvenue. Elle prévoit en outre d’exclure les grands projets d’envergure nationale et européenne des enveloppes foncières locales, qui ne viendront plus pénaliser le développement des territoires ; nous avons entendu avec tenus précédemment par M. le ministre à ce sujet. Enfin, elle renforce la place des élus locaux du bloc communal au sein de la conférence régionale du ZAN, portant leur représentation à 75 %. Ces ajustements sont nécessaires, mais sont ils suffisants ?

Pour assurer la prise en compte des spécificités locales, je crois également souhaitable de renforcer la représentation départementale au sein de la conférence régionale et d’éviter la mutualisation à l’échelle régionale du potentiel de développement des communes rurales, afin d’éviter son absorption par les zones urbaines. dit, l’enjeu le plus transversal reste la reconnaissance insuffisante de la diversité des territoires. Le recours à la grille de densité communale de l’Insee permettrait d’ajuster les règles aux réalités des territoires ruraux. Il ne peut y avoir une seule et même norme

secondé par quelques brillants éléments des élites de la technostructure et un bataillon de ministres redevables. Tout cela n’a eu qu’un temps et le sujet qui nous occupe aujourd’hui en est la plus parfaite illustration. En effet, la loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, était censée marquer un tournant décisif dans la politique environnementale française. Ce texte ambitieux visait à accélérer la transition écologique du pays en s’attaquant aux principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Des transports à l’agriculture, en passant par le logement et la consommation, rien ni personne ne pouvait échapper aux contours d’une société plus durable et résiliente face aux défis climatiques. Et voilà que l’on nous invente une machine infernale, un sommet de planification bien de chez nous, un Gosplan à la française. Évidemment, tout cela se conçoit et s’écrit sans concertation, dans quelques cénacles autorisés, où l’on a la science infuse, puisque nous autres sénateurs sommes des ignorants Évidemment, tout cela s’envisage sans aucune étude d’impact sérieuse et chiffrée, puisque nous sommes déjà entrés de plain pied dans le « quoi qu’il en coûte ». Pourtant, ce salmigondis de 305 articles impose, pour les années à venir, des changements profonds affectant brutalement le quotidien des Français, des entreprises et des collectivités. Au beau milieu de ce fatras, on a même introduit un objectif national de zéro artificialisation nette d’ici à 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de la consommation foncière d’ici à 2031. Entendons nous bien, si l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols est unanimement partagé, il pose avant tout une question de modèle culturel. De quelle façon voit on la France de demain ?

Nous ne voyons pas la France comme l’ineffable Mme Wargon, qui osait qualifier avec mépris les maisons individuelles de « non sens écologique, économique et social ». Le chaos politique dans lequel Le chaos politique dans lequel nous a plongés cette démarche solitaire, aveugle et technocratique nous contraint désormais à nous rendre à l’évidence : croire que la politique peut s’improviser est une idée fondamentalement fausse.

Cet ancien monde, Gérard Collomb – paix à son âme – en était l’une des incarnations, et vous étiez fort justement à ses côtés, monsieur le ministre, lorsqu’il s’est agi de dénoncer, par exemple, la loi sur le cumul des mandats, dont on mesure aujourd’hui les effets délétères. Souvenez vous de ses derniers mots – presque un règlement de compte – lorsqu’il a claqué la porte : il a mis en garde publiquement contre la déconnexion à l’égard des territoires. Aussi, monsieur le ministre, au regard de votre parcours, qui atteste merveilleusement de votre enracinement dans ces territoires de France, tempérez donc les ardeurs d’une administration devenue folle et laissez votre collègue Mme Pannier Runacher à son « saut quantique », dont on connaît l’issue.

Toutefois, cette définition reste trop restrictive et exclut de nombreux territoires dans lesquels l’urbanisation s’est historiquement développée sous forme de hameaux dispersés

L’incapacité des maires d’y autoriser des constructions freine le développement local, contribue à la rareté du foncier disponible et accentue la pression immobilière sur d’autres secteurs déjà saturés. Il est donc nécessaire d’adapter les critères définissant les secteurs déjà urbanisés, en reconnaissant la spécificité des hameaux comme partie intégrante du tissu communal, afin de permettre leur densification maîtrisée et d’offrir des solutions de logement adaptées aux besoins locaux. Cette évolution législative permettrait de résoudre des difficultés locales propres aux territoires à urbanisation diffuse, tout en garantissant une urbanisation cohérente et encadrée. À l’instar de la jurisprudence récente du Conseil d’État, qui a assoupli les critères de densité pour les secteurs déjà urbanisés, il conviendrait d’étendre cette approche aux hameaux, dès lors qu’ils disposent de voies de circulation, d’équipements et d’un raccordement aux réseaux publics. En reconnaissant ces espaces comme éligibles à une densification progressive, on éviterait une artificialisation excessive

En effet, il nous avait été signalé que les élus avaient du mal à appréhender cette notion pourtant essentielle pour appréhender celle de consommation d’Enaf. La définition de l’enveloppe urbaine correspond, de fait, à l’ensemble des espaces urbanisés en continuité, y compris les dents creuses.

au delà de la dernière construction reviendrait à favoriser l’extension urbaine, alors que votre préoccupation concernant les dents creuses est satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 1. Quant au sous amendement n° 184, il a pour objet de considérer que tout hameau constitue une enveloppe urbaine. Or cela ne doit pas être automatique : selon leur configuration, notamment leur densité, certains hameaux pourront être qualifiés d’espaces urbanisés, donc former une enveloppe urbaine, et d’autres non.

Céline Brulin, pour explication de vote.

la poursuite du projet urbain, la recherche de la sobriété foncière et la capacité à préserver les paysages, les habitats naturels et les fonctions productives des sols. Réduire l’artificialisation des sols à la seule consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers conduirait ainsi à méconnaître les dynamiques urbaines et de résidentialisation. L’article L. 371 1 du code de l’environnement précise d’ailleurs que les trames verte et bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu Ces corridors de conservation contribuent de manière significative à la résilience des paysages en favorisant la croissance de la végétation, la biodiversité et la présence les pollinisateurs naturels, qui profitent aussi à l’agriculture. À mesure que ces corridors s’étendent, ils deviennent de puissants puits de carbone, contribuant à atténuer les effets du changement climatique. Tel devrait être l’objectif, afin de ne pas faire de la désartificialisation des sols un totem, mais bien d’encourager la renaturation, lorsque cela est possible, en optimisant la recherche de corridors écologiques.

En effet, la mesure des espaces urbanisés se fait dans la maille de la subdivision fiscale, qui est plus petite, je le précise, que celle de la parcelle cadastrale. Or, bien que j’en comprenne l’intention, l’écriture proposée par la commission pose plusieurs difficultés.

l’amendement n° 163, exclure de la non comptabilisation de la consommation d’Enaf les parcelles en bordure d’enveloppe urbaine lorsqu’elles sont majoritairement entourées d’espaces bâtis ou lorsque le sol est déjà imperméabilisé semble contre productif.

Comment comptabiliser une parcelle composée d’un pavillon et d’un jardin ? Nous retomberions dans les difficultés de comptabilisation qui crispent les élus. Je vous demande donc, ma chère collègue,

C’est l’objet de l’amendement que le Gouvernement a déposé sur l’article 1 pour rétablir un faisceau d’indices à la fois lisible, sécurisant juridiquement et assez souple pour que les élus puissent

Chaque territoire doit pouvoir s’appuyer sur un faisceau d’indices tenant compte de caractéristiques spécifiques, telles que le type d’urbanisation, sa continuité, la quantité et la densité des constructions, la structuration par des voies de circulation ou par des réseaux ou encore la présence d’équipements. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens. Votre amendement va bien plus loin en fusionnant la notion d’espaces urbanisés avec celle de secteurs déjà urbanisés

hameaux intégrés à l’environnement » dans la définition de la consommation d’Enaf. Cet ajout aurait pour effet de complexifier inutilement la définition proposée. Le texte de la commission définit la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés. En pratique, cet amendement est donc déjà satisfait par la rédaction actuelle, raison pour laquelle j’y suis défavorable. L’amendement n° 163 vise à revenir sur la proposition de la commission, selon laquelle l’étalement urbain en bordure de l’enveloppe urbaine ne doit pas être comptabilisé comme une consommation d’Enaf.

Par ailleurs, la consommation d’espace peut avoir lieu à une échelle inférieure à celle de la parcelle. Les outils de mesure de la consommation de l’espace naturel mis à disposition par le Cerema sont d’ailleurs à une maille infraparcellaire.

De façon générale, le texte adopté en commission a pour ambition de faciliter l’intégration des constructions au sein de l’enveloppe urbaine, en considérant qu’il ne s’agit pas de consommation d’Enaf.

Néanmoins, tous les espaces interstitiels dans l’enveloppe urbaine ne se valent pas. La jurisprudence fait souvent valoir des critères de taille. Les petites parcelles sont par exemple considérées comme des dents creuses. La disposition que vous proposez

ou non. Je comprends l’intention d’apprécier différemment les surfaces imperméabilisées et les surfaces non bâties dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur un territoire.

établit une dichotomie stricte entre les surfaces artificialisées ou non, qui ne tient pas compte du potentiel de renaturation des sols construits. cet amendement, nous proposons d’établir par décret une nomenclature des sols artificialisés fondée sur un gradient d’artificialisation associé, pour chaque niveau, à un coefficient intégrant la qualité des sols. Cette nouvelle matrice permettrait une gestion des sols à la fois plus fine et plus flexible à l’échelle de chaque territoire.

des sols artificialisés n’a plus de sens. Au contraire, c’est pour échapper à cette nomenclature complexe et mal comprise des élus, qui nous a valu tant de débats avec les précédents gouvernements, que nous voulions en revenir aux Enaf, notion que les acteurs locaux connaissent et maîtrisent. Par conséquent, l’avis de

doublons. Vous le savez, le code général de l’urbanisme prévoit un suivi de la consommation foncière, qui doit être intégré au schéma de cohérence territoriale.

les Scot. En l’état actuel du droit, les Scot et les plans locaux d’urbanisme sont amenés à faire l’objet d’un double bilan de leur consommation foncière, car deux périodes s’imposent actuellement

qui n’est pas couvert par votre amendement, et maintenir le bilan sur les années précédant directement l’arrêt du projet pour permettre aux collectivités de tenir compte des coups partis. Je suis donc favorable à ces amendements et je proposerai d’élargir le dispositif aux PLU et PLUi lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

La séance est levée.